conduite par M. Titus Corlatean, président de la commission des affaires étrangères du Sénat roumain. La délégation est accompagnée de M. Bernard Fournier, président du groupe d'amitié France-Roumanie. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires réguliers qu'entretiennent les Sénats français et roumain, portera en particulier sur l'actualité européenne, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ainsi que sur la francophonie. Permettez-moi de souhaiter à nos amis roumains un séjour et des échanges fructueux, en formant le voeu que cette rencontre interparlementaire contribue à renforcer encore les liens d'amitié qui unissent nos deux assemblées. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Sénat français. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

madame la vice-présidente de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames, messieurs les sénateurs, nous y voici ! Après plus de huit mois d'intenses travaux, pour sonder les difficultés de l'institution judiciaire, et près d'un million de contributions citoyennes ; après la remise du rapport du comité des États généraux de la justice ; après deux grandes vagues de concertations, à l'été et à l'automne derniers, avec l'ensemble des parties prenantes du monde judiciaire ; après la présentation d'un plan d'action global pour la justice en janvier dernier ; après donc toutes ces étapes, nous voici réunis aujourd'hui pour discuter de la première traduction législative et organique de ce plan d'action. Conformément à l'engagement du Président de la République et de la Première ministre, je viens vous présenter les projets de loi de programmation et de réforme du statut de la magistrature les plus ambitieux de l'histoire du ministère de la justice. Pour vous parler très simplement, comme je l'avais fait sur le perron du ministère en juillet 2020, lors de mon entrée en fonctions, je viens surtout tourner, avec vous, la page des mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis plus de trente ans. La première de ces mauvaises habitudes est celle qui consiste à demander toujours plus à la justice, tout en lui donnant toujours moins. Oui, je suis venu tourner avec vous la page du délabrement, de la « clochardisation » de la justice française ! La route est encore longue, bien sûr, mais nous allons désormais dans la bonne direction, d'un pas résolument assuré.

de ces habitudes est sans doute la pire : ne pas placer au coeur des réformes le justiciable, qu'il soit victime, accusé, demandeur ou requérant. Je le dis clairement, avec ce plan d'action et ces projets de loi, nous avons pour ambition de répondre concrètement aux attentes de nos concitoyens,

Vous l'aurez compris, notre priorité absolue est de donner à la justice les moyens nécessaires pour lui permettre d'être à la hauteur de sa mission. C'est pourquoi, à l'article 1 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice, je vous propose d'entériner une hausse inédite des crédits de la justice, qui atteindront près de 11 milliards d'euros en 2027. Au cours des cinq prochaines années cumulées, les crédits du ministère de la justice augmenteront de près 7,5 milliards d'euros,

qui correspondent, de manière globale, aux enjeux d'efficacité du service public de la justice. Le premier objectif, la mère de toutes les batailles, c'est le recrutement massif et rapide de magistrats, de greffiers, d'attachés de justice, d'agents pénitentiaires et d'agents administratifs ; bref, de tous ceux qui font vivre le ministère de la justice. Pour graver cela dans le marbre, j'ai souhaité inscrire dans le

deuxième objectif est la revalorisation de ceux qui servent notre justice au quotidien. Pour recruter massivement, il faut attirer les talents vers le monde de la justice.

et des officiers de la catégorie B à la catégorie A. Il était grand temps de reconnaître le rôle indispensable de la troisième force de sécurité intérieure de notre pays ; je suis fier non seulement d'être leur ministre, mais surtout d'avoir amélioré leur place dans la fonction publique.

ils sont freinés par une informatique et un réseau qui ne sont pas à la hauteur. Le but est clair : comme dans la juridiction administrative, il faut instaurer le zéro papier à l'horizon 2027. Pour cela, nous avons une méthode. Nous dotons d'abord toutes les juridictions d'experts en informatique qui

Nous accélérons la mise à jour, concertée avec le terrain, des logiciels en matière civile ; je pense par exemple à Portalis. En matière pénale, ce projet de loi de programmation prévoit le déploiement, déjà engagé, de la procédure pénale numérique, en lien avec le ministère de l'intérieur. À cet effet, un chef de file unique sera issu de la Chancellerie. La transformation numérique de la justice doit également se faire en direction de ceux qu'elle sert, c'est-à-dire bien sûr des justiciables. En janvier dernier, j'annonçais le lancement d'une application sur smartphone regroupant des fonctionnalités importantes. C'est chose faite : elle a été lancée le 27 avril dernier dans une version qui permet déjà, par exemple, de savoir si, oui ou non,

d'abord, bien sûr, de l'immobilier judiciaire, c'est-à-dire de la construction de tribunaux. Les recrutements massifs vont nécessiter une augmentation et une rénovation massives du parc judiciaire. C'est pourquoi nous avons une vision et une stratégie globales : nous prévoyons d'investir de manière massive dans les tribunaux de demain afin d'agir sur tous les leviers d'amélioration des conditions de travail

de restructuration et de rénovation de tribunaux et de cours. Ensuite, il y a le programme immobilier pénitentiaire, qui avance sûrement, malgré les nombreux freins, comme la crise sanitaire- si elle est derrière nous, elle a durablement affecté les chantiers -, la guerre en Ukraine, qui a réduit l'accès aux matières premières, et, bien sûr, les réticences des riverains et, souvent, de leurs élus. Notre engagement est clair et notre cap est fixé : nous construirons 15 000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027. L'année prochaine, la moitié des établissements prévus dans ce plan seront sortis de terre. Il y va d'abord de la bonne application de ma politique pénale, qui est sans aucune ambiguïté : fermeté sans démagogie, humanisme sans angélisme. Il y va ensuite des conditions de détention, qui sont parfois indignes. Je fais le tour des prisons depuis plus de quarante ans, je connais la dégradation d'un certain nombre d'établissements, mais je n'ai pas de baguette magique : je n'ai qu'une volonté politique forte, des leviers d'actions réalistes et des moyens inédits. En matière pénitentiaire comme en matière pénale, il faut se méfier des solutions miracles, clés en main. La construction de prisons est la solution la plus lente, mais la plus sûre, d'autant que, en parallèle des constructions, nous investissons massivement dans les rénovations, pour un montant de près de 130 millions d'euros par an, soit près de deux fois plus que sous le quinquennat de François Hollande. de la justice, l'a indiqué en quelques mots : tout ne se résume pas à la question des moyens. C'est pourquoi je vous propose une série de mesures qui viennent réformer en profondeur l'institution sans pour autant la déstabiliser. Oui, l'une des innovations de ce projet de loi de réforme de la justice, c'est de mettre en face des réformes les moyens nécessaires pour les appliquer correctement. Le premier axe de la réforme est l'amélioration de l'organisation de la justice, selon une approche innovante et pragmatique. Je souhaite accélérer la déconcentration du ministère de la justice en laissant plus d'autonomie aux juridictions dans leur administration, afin de ne faire intervenir l'administration centrale que lorsqu'elle est utile en matière de support ou nécessaire en termes d'arbitrages. Il faut faire confiance aux acteurs de terrain

à ce projet de loi, car une organisation plus efficace de la justice, ce sont aussi des moyens mieux employés, au plus près des professionnels et des justiciables. L'amélioration de l'organisation des juridictions passe aussi par des expérimentations innovantes visant à améliorer concrètement le service rendu au justiciable. C'est ce que nous proposons, à travers l'expérimentation d'un véritable tribunal des activités économiques. En effet, l'organisation actuelle des juridictions commerciales manque de lisibilité pour les justiciables et les différents acteurs. Je vous propose également d'expérimenter une contribution économique, comme cela se pratique dans divers pays européens, afin notamment de lutter contre les recours abusifs

Je souhaite évidemment que tous les leviers à notre disposition soient employés pour nous assurer non seulement que le plan de recrutement sera réalisé, mais surtout qu'il correspondra aux besoins du terrain. Cette modernisation implique d'abord une adaptation des ressources de la Chancellerie à la réalité d'aujourd'hui, notamment celle de la diversification des fonctions. Je pense par exemple au travail formidable réalisé par les contractuels dans toutes nos juridictions. Leur recrutement, ainsi que l'engagement des magistrats et des greffiers,

30 %, c'est la moyenne nationale. Moins de stocks, c'est moins d'attente pour nos concitoyens ! C'est pourquoi, en plus des recrutements massifs

la possibilité de recruter des surveillants adjoints par la voie contractuelle. Cette approche a fait ses preuves au ministère de l'intérieur. J'ajoute que, en termes d'attractivité, le recrutement de contractuels permet d'embaucher des personnels au plus près des établissements pénitentiaires.

Recruter 1 500 magistrats va nécessiter de faciliter l'accès à la magistrature. Pour cela, nous proposons la création de magistrats en service extraordinaire, mais également une ouverture des recrutements, en simplifiant les différentes les différentes voies d'accès, notamment pour les avocats, et en professionnalisant le recrutement par l'instauration d'un jury professionnel. Le maintien du principe du concours républicain nous garantira évidemment l'excellence du niveau de recrutement. L'objectif est aussi d'assouplir

il convient également de simplifier certaines règles de gestion des ressources humaines. Je pense ainsi à la pérennisation des brigades de soutien de magistrats et de greffiers, qui ont récemment fait leurs preuves à Mayotte et en Guyane la mise en place des priorités d'affectation des magistrats qui ont accepté de partir dans des territoires peu attractifs ; ou encore, à la création d'un troisième grade, pour garder des magistrats d'expérience de

son dernier axe porte sur la responsabilité du corps judiciaire. Il s'agit notamment d'élargir à la fois les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables

Le troisième chantier de la réforme est la simplification d'un certain nombre de procédures : qu'elles soient civiles ou pénales, elles sont aujourd'hui un facteur de complexité pour nos professionnels et d'éloignement entre le citoyen et la justice. Vous le savez, en matière civile, je veux simplifier la procédure d'appel en réformant le décret Magendie et surtout faire enfin advenir la révolution de l'amiable, qui se fait tant attendre dans notre pays. Ces réformes relèvent du domaine réglementaire, mais j'ai transmis à la commission des lois le projet de décret concernant la mise en place de la césure et de l'audience de règlement amiable, afin que nous puissions échanger sur ces questions dans les semaines à venir,

le chantier titanesque de la simplification de la procédure pénale. Il s'agit, dans un premier temps, de restructurer

Pour garantir que cette réécriture se fera bien à droit constant, j'ai mis en place un comité scientifique et je vous proposerai, mesdames, messieurs les sénateurs, de créer également un comité de suivi composé d'un représentant par groupe parlementaire et des présidents

octroyée par le législateur. Par ailleurs, je vous confirme que le nouveau code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur avant la ratification de cette ordonnance, comme ce fut le cas pour le code de la justice pénale des mineurs et conformément à la volonté de votre commission et de ses rapporteures. Enfin, il vous est proposé une série de mesures concrètes immédiatement applicables. Je pense par exemple à des mesures améliorant l'efficacité de l'enquête pénale. Je pense également à l'extension des travaux d'intérêt général aux entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Je pense enfin enfin à l'extension du champ des infractions recevables pour une indemnisation des victimes. Pour conclure mon propos déjà trop long, je tiens à saluer le travail de la commission, de ses rapporteures et de son président. Si nous avons certaines divergences, sur lesquelles nous reviendrons lors de l'examen des amendements, je sais que nous partageons une ambition commune, en réponse à l'impérieuse nécessité de restaurer la place de la justice. à la hauteur de la mission fondamentale qui est la sienne, à la hauteur de l'engagement de ceux qui la servent et, surtout, à la hauteur des attentes des Français, au nom desquels, ne l'oublions jamais, la justice est rendue.

ce désamour pour le juge ni le malaise persistant des acteurs de la justice n'ont été endigués par les six réformes législatives votées depuis 2017, dont la dernière, baptisée « loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », date de moins d'un an et demi. L'enchevêtrement des réformes successives n'a pas résolu la crise que la justice traverse depuis plusieurs années. Comme le résume Jean-Marc Sauvé dans le rapport qu'il a remis à l'issue des États généraux de la justice, cette situation découle d'un « malaise profond » aux origines lointaines, que l'ordonnancement juridique actuel,

Toutefois, certaines dispositions restent très en deçà de l'ambition exprimée lors des États généraux de la justice. C'est le cas de la réforme du témoin assisté, ainsi que de la constitution de l'équipe autour du magistrat, équipe dont sont exclus les greffiers. Le chantier de la réforme de la justice n'est pas qu'une affaire comptable, même si les moyens ont leur importance. L'effort budgétaire, de 6,80 % à euros constants, inscrit dans la durée pour les années 2023 à 2027, est assurément bienvenu. Cela permettra notamment de financer les postes promis : 1 500 magistrats et 1 500 greffiers. Ces recrutements contribueront à combler notre retard par rapport à nos voisins européens. Nous avons souhaité augmenter l'ampleur des recrutements de greffiers, dont le rôle est central, et flécher 600 postes de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) afin de mieux accompagner l'exécution des peines. Mais ces moyens supplémentaires ne suffiront pas à atteindre l'objectif fixé sans une réforme en profondeur de l'organisation du travail des magistrats ni une véritable simplification des procédures applicables. Mes chers collègues, la réorganisation passe par une révision importante du corps judiciaire, corollaire des recrutements attendus. La commission des lois a souhaité d'abord ouvrir davantage le corps judiciaire, corps judiciaire, en prévoyant que les magistrats constitueraient moins de la moitié du nouveau jury professionnel, tout en renforçant le niveau d'exigence pour le recrutement et la formation de ces nouveaux magistrats.

Enfin, nous avons souhaité renforcer le pouvoir des chefs de cour d'appel, futures clés de voûte de la déconcentration des services judiciaires dans la gestion des ressources humaines, et ce dans le respect du principe d'inamovibilité des magistrats, corollaire de leur indépendance. En contrepartie, l'évaluation à 360 degrés des chefs de cour et de juridiction est alignée sur d'autres évaluations similaires pour la haute fonction publique. Il en est de même pour la responsabilité des magistrats judiciaires, consolidée grâce à une clarification de la faute disciplinaire et à un renforcement de l'échelle des sanctions. La modernisation de l'organisation du travail des magistrats impose avant tout une évaluation réelle de leur charge de travail, afin d'affecter les moyens en fonction des besoins. Véritable serpent de mer, cette évaluation était attendue pour la fin de 2022 ... Espérons qu'elle remontera bientôt à la surface Très attendue, l'équipe autour du magistrat est réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire aux attachés de justice et aux assistants spécialisés, les greffiers en étant de fait écartés. Cette conception est loin du modèle exposé dans le rapport de Dominique Lottin, repris par les États généraux. La sédimentation des réformes pèse aussi sur la qualité du travail judiciaire et sur la sécurisation des décisions de justice. La simplification du code de procédure pénale, qui compte 2 400 articles aujourd'hui, est unanimement souhaitée. qui soit l'occasion de poser les questions de fond sur l'instruction, sur l'unification des enquêtes, sur la place du parquet. La méthode de l'habilitation pour réécrire à droit constant le code de procédure pénale n'emporte pas l'adhésion naturelle du Sénat. D'une manière générale, la Haute Assemblée n'est jamais encline à se déposséder de son pouvoir normatif au profit du Gouvernement, sans être assurée d'en contrôler les effets lors de la ratification. L'habilitation sollicitée pose plusieurs questions : comment réécrire à droit constant un nouveau plan du code de procédure pénale sans en modifier le fond ? Comment le mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ? Comment le clarifier sans véritablement le simplifier ? À ces questions, À ces questions, votre réponse ne peut être qu'une étape du travail de la simplification de ce code. C'est pourquoi la commission des lois a souhaité repousser l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'une année afin de laisser le temps de la ratification. Elle proposera par ailleurs

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner deux textes portant réforme de notre justice.

le projet de loi organique. S'il est utile d'ouvrir la magistrature et d'augmenter le nombre de magistrats, nous devons aussi entendre la défiance régulièrement exprimée à l'égard de la justice, certains pensant les juges intouchables. Il est vrai que, au vu des résultats des saisines du Conseil supérieur de la magistrature - 3 324 saisines au cours des dix dernières années ; 88 jugées recevables ; 7 plaintes renvoyées, aucune sanction -, on pourrait le croire. L'indépendance de nos magistrats ne doit pas se confondre avec l'irresponsabilité. C'est pourquoi l'article 8 élargit les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables en supprimant la nécessité d'articuler les griefs. Articuler les griefs » : un juriste sait ce que c'est, mais pas un justiciable lambda. Or, sous le prétexte que l'on ne savait pas dire en droit quelle faute le juge avait commise, la demande était rejetée. Notre commission a également fait un choix de compromis en supprimant l'obligation d'audition systématique du magistrat, tout en clarifiant la définition de la faute disciplinaire et en renforçant l'échelle des sanctions. J'en viens à un sujet qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas : le niveau de diplôme requis pour exercer la profession d'avocat devient le master 2. Soit Mais le décret actuel qui définit les niveaux d'études requis ne distingue pas le niveau exigé pour exercer le métier de celui qui est requis pour intégrer le centre de formation. Or 8 % des élèves avocats n'ont qu'un master 1 et passent leur master 2 en cours de formation. Pourquoi se priver de ces élèves ? Il n'y a qu'un décret à changer pour distinguer les deux niveaux, monsieur

Sur ce sujet, nous avons fait le choix, avec ma collègue Agnès Canayer, de ne pas déposer d'amendements, en particulier sur le rapport annexé. Après tout, nous aurions pu faire

Pour le reste, ce texte porte une réforme de notre justice commerciale largement inspirée de l'excellent travail de nos collègues François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi. Nous expérimenterons donc des tribunaux des activités économiques. Pour autant, nous avons souhaité rendre cette réforme plus ambitieuse en l'étendant à tous les corps de métiers et en permettant à l'expérimentation de se faire dans les conditions réelles, avec des juges consulaires issus des différentes professions ajoutées. Autre point notable, l'instauration d'une contribution pour la justice économique : le Sénat y est favorable de longue date. Cette mesure figurait dans le rapport d'information de Philippe Bas de 2017, qui instaurait un droit de timbre pour responsabiliser les justiciables tout en finançant mieux la justice en général. sceaux, nous devons faire attention au montant de cette contribution, en particulier pour les acteurs économiques en difficulté. Si celle-ci est pertinente, elle ne doit pas devenir un frein à l'accès à notre justice.

dégradation de l'institution judiciaire », « souffrance du personnel de la justice », « incompréhension des justiciables» : ces mots sont issus du rapport du comité des États généraux de la justice de juillet 2022. Ce rapport appelait à une réforme systémique dans un contexte de défiance généralisée face aux institutions. Or les deux textes que nous examinons aujourd'hui ne répondent pas réellement à une telle ambition.

De même, nous restons dubitatifs sur la pratique du rapport annexé, qui permet de tout dire, mais qui n'a aucune valeur législative et qui peut être une manière de se défausser.

de ses mesures étant attentatoires aux libertés. Le renvoi de certaines procédures au juge des libertés et de la détention au motif d'alléger l'organisation des audiences et la charge des tribunaux correctionnels nous semble plutôt être une manière détournée de gérer les flux liés au nombre

Compte tenu des réserves qu'elle suscite, nous doutons de son intérêt. À tout le moins, nous estimons qu'elle n'est pas mûre en l'état. Enfin, le cadre d'action des nouveaux attachés de justice nous semble devoir être précisé,

de ne pas complètement déséquilibrer la composition du corps des magistrats. Il convient aussi de veiller à ce que la durée de formation, comme la question du stage probatoire, réponde bien à ces objectifs. Prenons garde à ce que cette ouverture ne soit

Enfin, concernant l'introduction du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous regrettons que le texte traduise le renoncement à appliquer l'article 56 de la loi Sauvadet de 2012, désormais codifié à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, pour les nominations aux plus hauts postes de la hiérarchie judiciaire.

Sur le fond, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 affiche l'objectif d'une justice plus rapide, plus claire, en somme d'une justice moderne. Nous partageons bien évidemment cet objectif, mais nous regrettons l'absence de dispositions ayant vocation à endiguer la surpopulation carcérale. le projet de loi ne prévoit que la construction de 15 000 places de prison d'ici à 2027, ce qui est clairement insatisfaisant à nos yeux. Malgré les demandes, les tribunes, les alertes, rien n'a été envisagé en matière de régulation carcérale rien non plus sur la qualité du suivi en milieu ouvert. L'assignation à résidence avec surveillance électronique est devenue l'alternative à l'incarcération, alors qu'elle reste contraignante, désocialisante et qu'elle ne constitue pas une solution pour la réinsertion.

judiciaire et ne peuvent constituer une solution à long terme. La justice est un service public exigeant, qui ne saurait se passer de véritables magistrats, formés aux fonctions difficiles qui sont les leurs.

qui préfèrent les fonctions juridictionnelles et n'ont pas d'appétence pour les fonctions d'encadrement ou de coordination de service, encore moins pour l'exercice professionnel au sein de la haute hiérarchie judiciaire.

Pourtant, c'est moins à l'ouverture vers l'extérieur qu'à la simplification des voies de recrutement, à l'amélioration de la formation, puis à l'intégration des magistrats nouvellement recrutés qu'il faut selon nous s'atteler. À cet égard, le texte comporte de maigres avancées. Nous souhaitons donc rappeler que la magistrature ne doit pas devenir demain une voie de repli. La philosophie et la pratique de la magistrature ne sont pas les mêmes que celles de l'avocature.

Vous souhaitez aller vers une évaluation à 360 degrés des magistrats, ce qui revient à poser la question de la gestion des ressources humaines,

du CSM, ou plus exactement les modalités de reconduction des personnes qualifiées, en prévoyant une reconduction par moitié. C'est là un sujet qui a toujours interpellé la commission des lois. Le CSM agissant par

serait limitée à six mois. En bref, je ne vois pas d'autre solution pour réécrire le code de procédure pénale que de passer par la voie de l'ordonnance, sous réserve de bien se mettre d'accord sur son objet. Notre groupe

Monsieur le président, monsieur le ministre des détenus, mes chers collègues, la parole est à la défense, à la défense du peuple français ! Les justiciables sont dans l'incompréhension face à l'augmentation de l'insécurité, première des injustices, car elle porte atteinte à leur intégrité, à leurs biens, chèrement acquis, et à leur dignité. Les délais de jugement augmentent, les courtes peines et les peines de substitution à la prison se multiplient, les places de prison manquent toujours : il y a 73 000 personnes incarcérées dans les prisons françaises pour 60 900 places ; parmi ces oui, mes chers collègues ! Le désengorgement des prisons- certaines atteignent 200 % de leur capacité d'accueil - passe très clairement par l'expulsion de ces étrangers, qui constituent 23 % de la population carcérale. Les citoyens français veulent qu'on leur rende la sécurité, en restaurant une justice ferme et efficace et en rétablissant l'ordre dans nos prisons, car, même en prison, la violence règne encore. De leur côté, les magistrats sont soit politisés, soit découragés. Parmi les syndiqués, 33 % appartiennent au syndicat de la magistrature, qui s'est récemment illustré en mettant de l'huile sur le feu à Mayotte. Ce même syndicat, qui préfère dresser des « murs des cons » plutôt que de construire des murs de prisons, incarne une politisation de la justice. Ses outrances, sous prétexte de liberté syndicale, portent atteinte à la séparation des pouvoirs et nuisent à la confiance des Français dans la justice. Les autres magistrats sont découragés et contraints à un laxisme par défaut. Ils rendent des décisions sous la contrainte du manque de places en prison. Pour remédier à ce problème, vous proposez dans votre texte des places supplémentaires. Or, dans ce domaine, vous n'avez même pas atteint 6 % des objectifs fixés pour 2022 lors du premier quinquennat : vous aviez promis 7 000 places en net, il n'y en a que 400 à mettre à votre crédit. Qui peut croire, dès lors, aux 15 000 places supplémentaires dans quatre De plus, la confiance du peuple français en la justice va continuer de reculer, car vous éloignez le peuple et la société civile des structures qui la composent, en intégrant des magistrats professionnels dans les nouveaux tribunaux des activités économiques au détriment des milieux économiques et en n'élargissant pas le corps électoral des juges consulaires aux agriculteurs.

contre l'avis de la mairie et du barreau. Monsieur le garde des sceaux, de nouveau, vous faites l'unanimité contre vous ! Enfin, après le structurel, parlons politique. Comment croire que les choses changent vraiment quand le garde des sceaux, après s'être autoproclamé « ministre des prisonniers », assume comme une fatalité français (OQTF) ne puissent pas être exécutées ? Quel aveu de faiblesse et quel signal désastreux envoyé aux trafiquants d'êtres humains et aux clandestins ! Cette justice à deux vitesses assumée consacre la loi du plus fort. Pour vous, Lola est donc une victime inévitable. Vous faites ainsi un bras d'honneur à sa famille et aux justiciables, victimes de la barbarie devenue quotidienne. Vous siégez dans cet hémicycle sur le banc des ministres, mais, dans les faits, vous avez déjà démissionné. Votre démission est l'une des causes de la « décivilisation », car oui, après les trois années que vous avez passées à la tête de la Chancellerie, la France est plus que jamais

dès qu'il est question de réformer la justice, il est facile d'énoncer une série de lieux communs tant il y a maintenant longtemps que l'institution se dégrade : manque de matériel, locaux inadaptés, souffrance du personnel, incompréhension des justiciables. C'est bien simple : nos juridictions tiennent pour beaucoup grâce à l'engagement, au courage et à l'abnégation des magistrats et des agents qui les accompagnent quotidiennement- il me paraît indispensable de les soutenir. Il faut évidemment souligner les efforts budgétaires qui sont consentis depuis plusieurs lois de finances et qui tendent à replacer petit à petit notre pays à un niveau acceptable. À cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que cette dynamique se poursuivra dans les exercices à venir. Mais chacun le sait ici, le problème de la justice n'est pas exclusivement un problème de moyens. C'est aussi celui d'une institution qui peine à convaincre nos concitoyens de son efficacité. son efficacité. Lorsque la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire avait été annoncée, nous avions nourri l'espoir qu'elle apporterait une partie des réponses à ces problématiques. Il est regrettable que, moins de deux ans après l'adoption de ce texte, il faille de nouveau se pencher sur ces questions fondamentales, d'autant qu'il est justement reproché au législateur de trop souvent réformer espérons donc, une nouvelle fois, que la future loi n'aura pas besoin d'être suivie d'une autre dans quelques dizaines de mois. Sans quoi, nous devrons encore faire le constat d'une forme d'échec dans nos méthodes de travail. Sur le fond, sur un grand nombre de mesures proposées, le groupe du RDSE ne voit pas de difficultés majeures. C'est en particulier le cas concernant la mise en avant de la peine de travail d'intérêt général, l'élargissement du champ des infractions ouvrant droit à indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ou encore la déjudiciarisation de la procédure de saisie

Au RDSE, nous sommes très attachés à ce que le débat et le travail législatifs n'aient pas lieu en dehors des hémicycles et qu'ils s'y conduisent pleinement quand cela est nécessaire. Mais il faut aussi être lucide. efficace pour un tel objectif et la proposition de nos rapporteures de retarder d'un an l'entrée en vigueur de l'ordonnance est un bon compromis. Il demeure que, si la réécriture se fait à droit constant, nous pouvons aussi craindre qu'elle ne soit que partiellement satisfaisante.

En revanche, nous réservons encore notre position sur certaines mesures qui nous paraissent risquées du point de vue des libertés et au sujet desquelles des professionnels de la justice nous ont alertés. Je pense en particulier à deux dispositions de l'article 3. La première prévoit l'assouplissement du recours aux moyens de télécommunication pour les interprètes pendant la garde à vue et la téléconsultation médicale en garde à vue. Nous regrettons ce développement de l'usage de la visioconférence, notamment dans les cas où les personnes sont en situation difficile. Le projet de loi consacré à l'immigration, bien qu'il ne soit plus inscrit à l'ordre du jour, allait déjà dans ce sens et nous y étions alors opposés. J'ai du mal à envisager qu'une interprétation ou une consultation médicale ne perde pas significativement en qualité dès lors qu'elle se fait un micro et une caméra. qui nous inquiète, c'est l'activation à distance des appareils connectés des suspects aux fins de géolocalisation et de captation d'images et de sons. Les moyens d'investigation doivent être adaptés aux besoins des enquêteurs, surtout lorsqu'il est question de la sécurité nationale et de crimes et délits particulièrement graves. Vous nous permettrez néanmoins d'être sensibles à certaines préoccupations partagées par une partie des professionnels de la justice. Je pense notamment aux avocats, qui s'interrogent sur l'impact d'une telle mesure au regard des impératifs de confidentialité qu'ils entretiennent avec leurs clients. Sur ces deux dispositions, nous serons attentifs aux arguments qui seront avancés en réponse à certains de nos amendements. Si notre groupe est plutôt favorable à ce projet de loi, notre position pourrait évoluer en fonction de la teneur de nos débats. Je dirai enfin un mot concernant le projet de loi organique. Dans l'ensemble, nous y sommes favorables, même si nous tenons tout de même à relayer ici les regrets d'une partie des professionnels, notamment ceux du Conseil national de la magistrature, qui a pris une position assez critique sur ce texte. Cela Cela étant, il y a un intérêt réel à rénover les voies d'accès à la magistrature en les simplifiant, tout comme nous voyons un intérêt à responsabiliser davantage les magistrats.

est donc inévitable. Elle doit concerner les magistrats, les moyens matériels de la justice, mais aussi les greffiers et tous ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne judiciaire. Alors certes, le texte qui nous est soumis aujourd'hui a le mérite de répondre à des ambitions financières datant de depuis plusieurs décennies.

mais force est de constater que ces textes sont une réforme de l'institution judiciaire, alors que notre pays attend également une réforme en profondeur de la justice.

Or, face à la montée des violences dans notre pays, face au sentiment d'impunité qui explose, face aux zones de non-droit qui prolifèrent dans les cités, la France a besoin d'une révolution pénale. Sans cela, le ministre de l'intérieur, malgré son action résolue pour lutter contre l'insécurité, sera condamné, avec ses services, à vider la mer des délits et des crimes avec une petite cuillère percée. Cette révolution pénale passe avant tout par la construction de places de prison. C'est la seule garantie d'une bonne exécution des peines, la seule voie pour redonner du sens à la sanction pénale et mettre fin au sentiment d'impunité. Or ce projet de loi ordinaire prévoit des alternatives à la prison, comme la généralisation du recours aux travaux d'intérêt général et l'usage renforcé du bracelet électronique. Alors qu'il faudrait revenir sur les aménagements de peine pour rendre

les prisons et de 140 % dans les maisons d'arrêt, soit 73 000 détenus pour 60 000 places, faisant de la France l'un des pires élèves du Conseil de l'Europe en termes de surpopulation carcérale.

Pourtant, le président Macron avait promis 15 000 places supplémentaires d'ici à 2022. Au terme du premier quinquennat, on dénombrait seulement 2 000 places de prison supplémentaires

Il faut mettre en oeuvre des solutions incitatives afin d'encourager les communes à accepter davantage de tels projets. À cet égard, permettez-moi de vous livrer deux pistes de réflexion : la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement des communes qui se porteraient candidates à la construction de bâtiments carcéraux sur leur territoire

finir un dernier point : les ordonnances. Tout le monde s'accorde sur un point : il faut réformer le code de procédure pénale. Malheureusement, ce n'est pas ce que prévoit ce texte, sauf à la marge.

Sur ce sujet, les textes de loi comptent autant que les mentalités, parce que la justice est rendue par des êtres humains sur des affaires d'êtres humains. Il nous faut donc rechercher une adhésion large. À cet effet, chacun doit pouvoir dire sa vérité. Depuis trop longtemps, on a coupé la justice du peuple, en la laissant vivre en vase clos, en ne lui permettant pas de juger rapidement, en cultivant son incroyable complexité et parfois en minorant ses responsabilités. La justice retrouvera la confiance de tous les Français si elle permet de garantir leur sécurité, première des libertés. La

il structure désormais la plupart de nos sociétés. Rappelons-le, nous croyons aux vertus de l'État de droit. Nous croyons qu'il est bon que les droits et les devoirs soient démocratiquement définis. Nous croyons qu'il est nécessaire de respecter les libertés individuelles et la propriété privée. La confiance des individus dans l'institution judiciaire est un pilier indispensable au bon fonctionnement de la société. Or nous constatons qu'un doute s'est installé, qu'un fossé s'est creusé, puisque près d'un Français sur deux estime que la justice fonctionne mal. était l'objet du texte dont nous avons débattu il y a quelques mois. Depuis de nombreuses années, monsieur le garde des sceaux, votre ministère souffre d'un mal chronique. Il ne faisait pas partie des priorités politiques des gouvernements qui se sont succédé. Comme trop souvent, le long terme a été hypothéqué au profit de contingences immédiates. Or, lorsque la justice est délaissée, ce sont nos concitoyens et de nos entreprises qui en subissent les conséquences, c'est le pacte républicain qui se fissure. La question des moyens, à cet égard, est fondamentale. La France figure parmi les pays développés qui investissent le moins dans la justice : en 2020, notre pays y consacrait 72 euros par habitant, contre 111 euros au Royaume-Uni et 140 euros en Allemagne, soit le double

L'augmentation des moyens permettra la création de nouvelles places. Si les juges condamnent, les moyens pour que les peines soient bien appliquées font encore défaut. et de programmation doit également permettre de réduire les délais de jugement- vous avez parlé de les diviser par deux -et d'améliorer les conditions de travail dans les juridictions. Pour ce faire, il faut recruter plus de magistrats et veiller à l'attractivité de leur métier.

Si le manque de moyens explique beaucoup des difficultés auxquelles la justice fait face, ce n'en est pas la seule cause. La France compte environ quatre-vingts codes juridiques. L'inflation normative rend notre droit illisible et en partie impraticable. Le code de procédure pénale a triplé de volume depuis sa création.

Il nous semble qu'il sera nécessaire à cet égard de trancher une question qui revient souvent : la fusion des cadres d'enquête. La complexité actuelle nuit au travail des professionnels et aux droits de nos concitoyens. concerne les libertés individuelles, nous comprenons les inquiétudes légitimes que suscite le développement de techniques d'enquête de plus en plus intrusives, notamment l'activation à distance des micros et des caméras des téléphones ou des ordinateurs ou encore leur géolocalisation. Il est nécessaire de veiller à leur strict encadrement ; nous soutenons donc les dispositions qui interdisent leur utilisation dès qu'il est question de journalistes, de magistrats ou encore, pour ne pas dire surtout, d'avocats. Si le volet pénal est une composante essentielle de la justice, cette dernière englobe bien d'autres domaines. Nous soutenons l'expérimentation des tribunaux des activités économiques et il nous paraît cohérent que ces derniers soient chargés de l'ensemble des procédures relatives aux entreprises en difficulté. La commission a clarifié la composition de ces juridictions expérimentales ; c'était nécessaire et attendu sur le terrain. Autre innovation apportée par le texte : les saisies de rémunérations seront confiées aux commissaires de justice, sous le contrôle des juges.

mais plus que sur son montant, c'est sur sa répartition et sur son utilisation que nous nous interrogeons. En premier lieu, nous regrettons une fois de plus le « tout carcéral » que ces textes portent.

de prison supplémentaires n'est pas le seul remède. La punition d'exclusion sociale ne peut pas être découplée de l'objectif de réinsertion ; la situation des services pénitentiaires d'insertion et de probation en est un exemple. Notre pays a tout autant été condamné en raison de la surpopulation carcérale structurelle que pour l'absence de recours effectif permettant à un détenu de faire cesser des conditions de détention qu'un tribunal jugerait indignes.

Notre groupe a toujours défendu un système de justice équilibré et des mesures de privation de libertés encadrées. C'est pourquoi nous demanderons que soient étendus les droits de visite des parlementaires au sein des hôpitaux psychiatriques.

risque d'être contre-productive si celle-ci ne s'accompagne pas du maintien des démarches papier. Je l'ai dit à l'occasion de l'examen de nombreux textes : 13 millions de Français souffrent d'illectronisme à ce jour, et le tout internet ou le tout application peut dégrader leur accès au service public.

les deux textes que nous nous apprêtons à examiner en discussion commune sont le fruit de travaux menés au cours des États généraux de la justice, lancés en octobre 2021 à Poitiers par le Président de la République, et dont les conclusions, remises en juillet 2022, figurent dans le rapport Sauvé. Ils sont, en outre, la concrétisation législative d'une grande partie des soixante mesures du plan d'action, lui-même issu de ces États généraux,

de m'excuser, monsieur le garde des sceaux, mais je commence à être à court d'adjectifs pour saluer et caractériser l'augmentation de ces crédits ! Nous ne nous en plaindrons évidemment pas, car ces moyens financiers importants viendront renforcer les moyens humains indispensables au bon fonctionnement de cette institution et permettront de poursuivre tout à la fois le recrutement de personnels supplémentaires et la revalorisation des rémunérations et des carrières. Ce sont donc 10 000 personnes qui seront recrutées d'ici à 2027, dont 1 500 magistrats

La réforme statutaire, que nous examinerons concomitamment, vise à accompagner cette augmentation importante des effectifs de magistrats prévue par le projet de loi d'orientation et de programmation. Elle s'inspire elle aussi des recommandations formulées par le comité des États généraux de la justice et prévoit notamment d'ouvrir le corps judiciaire sur l'extérieur, d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats et le dialogue social, de développer la responsabilisation des magistrats et de renforcer leur protection. En outre, ces nouveaux moyens financeront la transformation numérique, ainsi que les chantiers immobiliers du ministère. J'entends les réticences concernant la construction de 15 000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027, mais je souligne que ces places sont nécessaires construction s'accompagne de mesures d'aménagement de peines, telles que l'extension du champ des travaux d'intérêt général ou encore de la libération sous contrainte. garde des sceaux, vous entendez également rationaliser l'organisation judiciaire et la répartition des contentieux entre les juridictions. À cet égard, je ne puis que me réjouir de la reprise, à titre expérimental, du tribunal des activités économiques, dont nous avions proposé la création, François Bonhomme et moi-même, dans une proposition de loi ratifiant, modifiant et complétant l'ordonnance

La commission a adopté deux amendements déposés par mon groupe visant à prévoir que le Parlement sera associé à l'évaluation de l'expérimentation des tribunaux des activités économiques et de la contribution pour la justice économique, ce dont je me félicite. Dans ce même esprit de rationalisation, vous proposez de procéder, par voie d'ordonnance, à la réécriture à droit constant de la partie législative du code de procédure pénale. Au comité scientifique, installé en janvier dernier, et composé de professionnels du droit, chargé d'assurer le suivi des travaux de réécriture, un contrôle parlementaire sera ajouté, afin de veiller à la conformité de la refonte du code de procédure pénale aux conditions et orientations de l'habilitation. Nous avons souvent débattu de l'idée selon laquelle les prérogatives du Parlement seraient mises à mal par le recours aux ordonnances lors de l'examen de textes d'habilitation. Soyons honnêtes, il est assez inédit qu'un gouvernement mette en place une telle concertation

En avril dernier, le Sénat avait organisé, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, un débat sur l'état de la justice dans les outre-mer.

En effet, entre particularismes géographiques, pauvreté, fracture numérique, barrières linguistiques, défaut d'attractivité et insécurité, les outre-mer cumulent les difficultés en matière de justice.

Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous préciser comment ces recrutements massifs seront ventilés outre-mer et de nous communiquer l'état d'avancement des chantiers immobiliers. Vous vous êtes récemment rendus aux Antilles, où vous avez annoncé que, en Guadeloupe, les travaux de rénovation de l'ancien palais, qui accueillera le conseil des prud'hommes, vous avez indiqué que la livraison d'une structure d'accompagnement vers la sortie interviendrait au premier trimestre 2025. À Mayotte, lors de votre déplacement en mars 2022, vous aviez annoncé la création d'une nouvelle cité judiciaire, d'un second centre pénitentiaire et d'un centre éducatif fermé. La réalisation de tels projets prend certes d'autant que nous faisons face à un énorme problème de foncier, mais il me semble important, compte tenu des événements qui frappent ce département, qu'un calendrier de mise en oeuvre puisse être rapidement dévoilé. En tout état de cause, et nonobstant les effets de tribune de certains, qui apparaissent finalement en décalage avec l'esprit constructif qui a présidé à l'examen de ces textes en commission, le groupe RDPI considère, pour sa part, qu'ils mettent en place une stratégie globale et à long terme pour moderniser notre système judiciaire. Le Gouvernement a pris la mesure des défis auxquels l'institution judiciaire est confrontée, tels que la surpopulation carcérale, les délais de procédure excessifs

voilà dix ans exactement, le Sénat votait à l'unanimité une proposition de loi que j'avais déposée visant la compétence universelle du juge français pour les infractions et les crimes relevant de la Cour pénale internationale

ressortissant. À cet égard, certaines décisions ont été prises, y compris par la Cour de cassation, qui ont suscité une réprobation internationale, comme vous le savez. Le 12 mai dernier, la Cour de cassation a pris une position claire sur la double incrimination,

Les constats effectués dans ce rapport, je ne vous apprends rien, étaient alarmants : difficultés dans l'exécution des peines, défaillance de l'administration pénitentiaire, délais de jugements toujours plus longs, etc. Cette situation est principalement due au manque de moyens alloués à la justice. Dès lors, les projets de loi que nous étudions aujourd'hui sont les bienvenus. qu'ils ouvrent, s'ils sont de bon augure, ne permettront pas, à eux seuls, de pallier les carences dénoncées dans le rapport Sauvé. Pour ma part, j'évoquerai simplement quelques aspects du projet de loi d'orientation et de programmation.

il s'agit de revenir sur les règles particulièrement sensibles touchant aux libertés individuelles et au pouvoir coercitif de l'État, lesquelles me paraissent relever beaucoup plus du législateur que du Gouvernement.

Et il ne faut pas oublier le flottement jurisprudentiel qui entoure la ratification de ces ordonnances. Je ne suis donc pas favorable à la méthode qui a été retenue. Sur le fond, ce même texte contient des mesures qui réforment profondément les règles de la procédure pénale. On est loin de la réforme à droit constant annoncée. Tel est

On peut se poser de légitimes questions sur certaines des mesures proposées, comme l'activation à distance des appareils électroniques dans le cadre d'une enquête judiciaire. Il n'est pas conforme à nos usages de mettre en place des pratiques qui relèvent plutôt de régimes politiques totalitaires

un magistrat du siège en qualité d'assesseur, qui serait désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce recours au principe de l'échevinage dans le tribunal des activités économiques est particulièrement mal perçu par les juges consulaires, qui y voient un signe de défiance, alors que les tribunaux de commerce ont su s'organiser pour rendre une justice dont la qualité n'est pas contestée. Le risque est grand, si cette disposition est maintenue, de provoquer une vague de démissions chez les magistrats consulaires alors que les tribunaux de commerce manquent aujourd'hui de juges. La commission des lois du Sénat l'a bien compris : elle a purement et simplement supprimé cette modification de la composition du tribunal des activités économiques. L'article 7 permet de déroger au principe de gratuité de la justice en instaurant une cotisation financière des entreprises, à la charge du demandeur devant le tribunal des activités économiques. Cet article, qui prévoit une mesure expérimentale dans certains tribunaux seulement, va créer une inégalité territoriale et ainsi entraîner, selon moi, une rupture d'égalité entre les justiciables. Il est également susceptible de porter atteinte à l'accès au droit pour les demandeurs de bonne foi qui devront, pour obtenir un titre de créance, payer non seulement cette contribution, mais aussi un avocat. Surtout, le fait de créer cette contribution constitue une première atteinte, notable, au principe de la gratuité de la justice, qui est la règle dans notre pays. Cette mesure n'est donc pas souhaitable. En résumé, la densité des observations qui sont faites à l'occasion de cette discussion générale montre, s'il en est encore besoin, l'importance et la complexité des deux textes concernés, tant sur la forme que sur le fond. Ce texte doit donc être modifié par notre assemblée, en ayant le souci non

pour mettre le droit et le fonctionnement de la justice au service de la lutte, prioritaire, contre les violences faites aux femmes ? Car,

Le rapport Sauvé, remis au garde des sceaux le 8 juillet 2022 et duquel découlent ces projets de loi, pointait particulièrement deux responsables de la crise que nous traversons : la sous-dotation permanente de l'institution judiciaire, ainsi que la complexification et la multiplication du droit et des procédures.

Chacun de ces tribunaux présente des problèmes structurels qui affectent l'efficacité de notre système judiciaire : manque de personnel, manque de moyens et défaillance, voire obsolescence, du matériel informatique.

Parmi ces objectifs figure la création de 15 000 places de prisons entre 2018 et 2027, pour lutter contre la surpopulation chronique dans ces établissements. Nos maisons d'arrêt présentent un taux d'occupation moyen de 143 %. Des milliers de places supplémentaires seraient nécessaires dès aujourd'hui pour que nos détenus soient accueillis dans des conditions acceptables.

Il dénonce le retard que prend l'exécution des programmes déjà lancés : seuls 35 % des 7 000 places annoncées en 2018 ont effectivement été mises en service et tout porte à croire que le délai ne sera pas tenu. Ces places sont pourtant indispensables pour que nos tribunaux puissent réellement remplir leur office et condamner nos délinquants à des peines effectives. À Bordeaux, les magistrats m'ont fait part d'une réalité aberrante : les prévenus ne sont plus condamnés à des peines de prison ferme afin de ne pas accroître la surpopulation carcérale du centre de Gradignan

Pour conclure, ces textes ne constituent malheureusement qu'une traduction approximative des recommandations évoquées précédemment. En effet, s'ils comportent des avancées réelles, comme le recours accru aux travaux d'intérêt général et l'expérimentation, réclamée de longue date

en portant par exemple l'objectif de recrutement de greffiers à 1 800 postes, mais l'écueil principal de cette réforme demeure. En procédant à une refonte par ordonnances de la procédure pénale, quelle place le pouvoir exécutif laisse-t-il au législateur pour réformer des règles extrêmement sensibles, qui touchent aux libertés individuelles et aux pouvoirs coercitifs de l'État ? ? Il est indispensable que le Parlement puisse contrôler le respect du champ de l'habilitation qu'il accorde au Gouvernement et qu'il dispose, surtout, du temps nécessaire pour le faire dans des conditions sereines.

Cette répartition sera fonction, bien sûr, des besoins des métiers, de l'avancement des projets, des capacités de recrutement, de la formation et des écoles.

Je n'ignore rien du rôle qu'ils jouent dans les juridictions. Je le redis, ils feront partie de l'équipe autour du magistrat. Ils sont indispensables aussi pour l'accueil des justiciables.

qu'il nous faut recruter de nombreux magistrats, que si les magistrats de l'ordre administratif souhaitaient venir abonder l'ordre judiciaire, il était tout de même normal qu'ils perçoivent le même salaire.

avec d'autres concours d'accès à des professions juridiques, notamment l'École nationale de la magistrature (ENM), qui, elle, ne fixe pas de limites quant au nombre de tentatives autorisées. Nous soutenons donc qu'il est essentiel de garantir l'égalité des chances et l'accessibilité à la profession d'avocat.

Enfin, il existe un numéro d'accès au droit, le 3039, qui reçoit environ 500 appels par jour.

Est-ce à dire que les amendements que nous allons examiner ne pourront être adoptés que si le Gouvernement y est favorable,

au moment où je vous parle, un suivi psychiatrique est préconisé pour la moitié des entrants en prison. Un sur deux ! Nous avons salué la création de nouvelles UHSA, mais nous souhaitons

pour déterminer les moyens réels, en développement et en construction, nécessaires à la prise en charge de détenus souffrant de difficultés psychiatriques.

les deux tiers des hommes et les trois quarts des femmes sortant de prison ont au moins un trouble psychiatrique ou lié à l'usage de stupéfiants. La seconde est en cours et s'achèvera en 2024 : elle vise également à évaluer la santé mentale des personnes incarcérées en maison d'arrêt.

que trois nouvelles UHSA seront prochainement construites en Île-de-France, en Normandie et en Occitanie, et que les établissements publics de santé mentale seront sécurisés, particulièrement en outre-mer.

en provoquant un engorgement des affaires en cours, ce qui a engendré une accumulation des dossiers en attente. Le délai impératif imposé par ce décret, sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, a contribué à cette situation.

et garantir ainsi des décisions de meilleure qualité.

vous indiquiez lors de la rentrée solennelle du barreau de Paris que, la semaine suivante, vous présenteriez une réforme de l'ordre de la procédure civile et de la procédure pénale, notamment celle du décret Magendie.

Cette simplification doit permettre la sécurisation juridique, la recherche d'une plus grande efficacité, l'allégement du poids des contraintes formelles, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement. Un comité scientifique composé de professionnels du droit de tous horizons sera chargé de formuler des propositions de clarification du code qui serviront de base à cette ordonnance de recodification à droit constant prévue à l'article 2, qui lui-même vise à engager la simplification attendue.

nous souhaitons que les travaux de réforme du code de procédure pénale pendant cette période soient limités pour assurer une stabilité attendue par tous les acteurs du monde de la justice. L'amendement n° 159, présenté

le développement de procédures de jugement rapide, en particulier la comparution immédiate, est pourvoyeur dans l'immédiat d'un plus grand nombre d'incarcérations et aboutit à un taux plus important de peines de prison ferme et à des peines plus longues. Pour l'instant, rien ne démontre si c'est le cas ou non. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y aurait un rapport mécanique entre la multiplication des procédures de comparution immédiate et la hausse du nombre de personnes incarcérées.

J'ai toujours affirmé que la méthode que nous choisissions pour clarifier un certain nombre de règles

par la rapporteure concernant l'organisation des travaux de recodification du code de procédure pénale, ce qui est important- j'espère que c'est bien comme cela qu'il faut entendre le propos tenu à l'instant par le garde des sceaux -c'est la phrase : « Lui seront présentés tous les trois mois l'état de leur avancement et les propositions de clarification et de simplification ... » Nous aurons largement l'occasion de débattre tout à l'heure

Mme la rapporteure

si, dans l'amendement qui a été voté à l'instant figure effectivement la création d'un comité de suivi et d'évaluation, c'est parfait. Je retire mon amendement.

important de comportements du fait de la création de nouveaux délits systématiquement assortis de peines d'emprisonnement ou du fait de l'aggravation de peines d'emprisonnement qui existent déjà. Ces derniers mois, plus d'une dizaine de textes de loi pénalisant de nouveaux comportements et durcissant les peines encourues ont été présentés et discutés au Parlement.

nous parlions. Notre groupe milite pour une meilleure individualisation des peines et pour une réponse pénale graduée, en évitant le plus possible l'incarcération en cas de courtes peines et en privilégiant pour ces dernières des mesures non carcérales, notamment par des mesures de probation en milieu ouvert. Quel est l'avis de la commission madame la rapporteure,

la mobilité de celui qui vient d'être condamné. Pourtant, je l'ai dit, ces travaux sont de moins en moins utilisés. Je demande dans toutes les circulaires que je prends qu'ils le soient davantage en précisant toujours- la précision est importante,

de prison. Vous parlez de limiter les possibilités de recours à la détention provisoire. Les dernières lois que je viens d'évoquer et l'article 3 du présent projet, que nous aborderons dans un instant, comportent des dispositions qui vont dans ce sens puisque nous souhaitons développer l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Dans la dernière circulaire de politique pénale que j'ai prise, le 20 septembre 2022, j'ai demandé que l'ensemble- je dis bien « l'ensemble » -de ces mécanismes

un processus spécialisé qui permet que les enfants n'aient pas à éventuellement témoigner plusieurs fois devant le père violent. C'est ce que je propose dans cet amendement : s'inspirer réellement du modèle espagnol

à M. Guy Benarroche. Le travail est l'un des moteurs de la réinsertion des détenus, mais l'exercice de cette activité en détention reste problématique malgré un certain nombre d'avancées récentes et au-delà des contraintes liées au milieu carcéral. Sur la question de la rémunération, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a récemment conclu à la non-conformité de la situation française avec le droit à une rémunération décente pour les personnes détenues, le paiement à la pièce, pièce, officiellement interdit, ayant toujours cours dans certains lieux. Dans les ateliers de production, le minimum légal est de 45 % du Smic, mais lorsque l'activité de travail concerne le bon fonctionnement de la prison, comme le nettoyage ou la cuisine, il oscille entre 20 % et 33 % du Smic.

en mesurer totalement les effets. Par conséquent, les évolutions que vous proposez sont peut-être à envisager, mais ultérieurement, lorsqu'un bilan de cette loi aura pu être dressé.

? Je suis d'autant plus défavorable à cet amendement, monsieur le sénateur, que le contrat d'emploi pénitentiaire qui a été voté il y a assez peu de temps, comme

Ils ne sont plus payés à la pièce : la pratique a totalement disparu. La France fixe des minimums de rémunération qui sont parmi les plus élevés

le détenu est tenu de rembourser ses victimes. Ce contrat d'emploi pénitentiaire est donc au moins triplement vertueux. D'abord, il y a sûrement à la clé un travail ou une formation, qui va dans le bon sens pour une réinsertion et pour l'absence de récidive. Ensuite, c'est intéressant pour les patrons : il y a un intérêt économique, mais également un engagement citoyen qui est fort. C'est enfin intéressant pour les victimes. le détenu a un certain nombre de droits sociaux : assurance chômage, assurance vieillesse, ouverture de droits en matière d'accident de travail, etc. Tout cela n'existait pas autrefois. Il s'agit donc là d'améliorations. Je pense que le travail est l'un des leviers qui permettent de lutter sérieusement contre la récidive. Le sens de l'effort n'est pas un sens interdit, ni en prison ni ailleurs. prison ni ailleurs. Avec ce contrat d'emploi pénitentiaire, nous ferons venir de plus en plus de patrons dans les établissements pénitentiaires pour fournir du travail.

Par ailleurs, la loi du 25 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur permet à toute victime d'une infraction pénale de déposer plainte.

Le ministère de l'intérieur prépare des décrets, notamment sur la question de la plainte par télécommunication audiovisuelle. À À ma connaissance, les Français se trouvant à l'étranger ne sont pas exclus de ce dispositif.

Aujourd'hui, la prise en charge totale des frais de justice s'applique à un revenu fiscal annuel inférieur à 11 200 euros, soit 938,50 euros par mois. Nombreux sont ceux qui ont un revenu légèrement supérieur, bien que très inférieur au seuil acceptable.

le rapport de la mission Perben relative à l'avenir de la profession d'avocat soulignait que le budget de l'aide juridictionnelle français se situait dans la moyenne basse de l'Union européenne et devait être rehaussé. Même si nous saluons la progression de 4,2 % des crédits budgétaires

est notamment due à la hausse du montant de l'unité de valeur, qui a dépassé en 2022, pour la première fois, son niveau d'origine en valeur réelle, c'est-à-dire corrigée de l'inflation.

je monte dedans avec mes amendements. Je vous suggère de faire de même, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à vos recommandations ! J'imagine par ailleurs que

: La parole est à M. Jean-Claude Requier. Le rapport annexé à ce projet de loi nous informe de la mise en place d'une application mobile à destination du citoyen et d'un site internet rénové. C'est une bonne chose pour permettre le développement du service public de la justice et faciliter son accès. Personne ne s'y oppose, même si nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'une priorité pour nos juridictions et les justiciables. Surtout, ces mesures ne doivent pas participer de la fracture numérique qui s'institue depuis plusieurs années. Le groupe du RDSE alerte sur ce risque régulièrement. Je pense en particulier au rapport qu'avait rendu notre collègue Raymond Vall. Il avait très bien souligné que, parallèlement à l'exclusion numérique diffuse que constitue l'illectronisme, il existe des exclusions numériques propres à certains publics tels que les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes sans abri, les personnes privées de liberté, ou encore les migrants. L'objet de cet amendement est donc d'indiquer que les innovations numériques liées au service public de la justice devront être accompagnées par des dispositifs luttant contre l'illectronisme. madame la rapporteure,

Requier, que le ministère de la justice s'intéresse à ceux de nos compatriotes qui n'ont pas accès aux nouveaux dispositifs numériques. Oui, c'est un sujet essentiel et nous sommes très vigilants sur ces questions.

la disponibilité en quantité suffisante de bracelets anti-rapprochement. Au lendemain d'un féminicide à Mérignac par un homme qui ne portait pas de bracelet, la presse avait révélé l'inégale répartition des bracelets anti-rapprochement entre les juridictions.

Le volume total de matériel ne cesse d'augmenter ; il sera porté en 2024 à 2 500 équipements. S'il en fallait davantage, nous en mettrions d'autres

quant à l'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre, par voie d'ordonnance, des mesures de clarification du code de procédure pénale. En effet, nous considérons que cette habilitation manque d'encadrement. Nous estimons qu'il est nécessaire d'aborder la rédaction d'un nouveau code de procédure pénale avec rigueur, temps et contrôle. Cette tâche complexe demande une analyse approfondie, la prise en compte des différentes implications juridiques, ainsi que l'écoute des experts et des acteurs du système judiciaire. Une approche précipitée ou insuffisamment réfléchie pourrait entraîner des lacunes ou des erreurs dans le nouveau code, compromettant ainsi son efficacité et sa cohérence. Aussi, nous considérons que le délai d'entrée en vigueur d'un an, tel qu'énoncé dans l'habilitation, est insuffisant.

à cet amendement.

à la fois les mentions du casier judiciaire et les mentions de restriction d'accès à certaines données dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Il s'agit ainsi de préciser que la mention inscrite dans le traitement d'antécédents judiciaires porte sur l'accessibilité des données, qui reste possible pour l'autorité judiciaire, mais qui n'est pas possible dans un cadre administratif.

La séance est suspendue.